Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie mardi 18 décembre sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.-

je vous propose, en accord avec le président et le rapporteur général de la commission des finances, de repousser le délai limite de dépôt des amendements, initialement fixé au début de la discussion générale, à la fin de celle-ci. Il

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes ici réunis pour examiner, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2019, compte tenu des désaccords manifestes entre les deux chambres. Après plus de 150 heures de débat au Sénat depuis sa présentation, je tiens à saluer votre implication et votre travail : vous avez déposé près de 2 000 amendements, introduit 101 articles et adopté 120 articles conformes

Cette nouvelle lecture est également l'occasion pour moi de revenir sur les annonces du Président de la République, qui répondent à l'urgence économique et sociale du pays. Ces annonces se sont d'abord matérialisées par la revalorisation de la prime d'activité, que vous avez adoptée à l'unanimité

retraités, qui font l'objet d'un texte que votre assemblée étudiera cette semaine. Bien que les modifications apportées par l'Assemblée nationale aient fait apparaître des divergences de fond évidentes entre la majorité présidentielle et la majorité sénatoriale, certains points de convergence méritent cependant d'être soulignés. S'agissant de l'impôt sur les sociétés, le Sénat a adopté conforme un article modifiant les règles de calcul des acomptes afin de permettre de mieux répartir les quotités d'impôt sur les sociétés dues par les entreprises. De la même manière, les deux chambres ont adopté sans modification l'article 17, visant à faciliter la croissance des entreprises en leur proposant un dispositif de révocabilité de leur passage de l'imposition sur les revenus à l'imposition sur les sociétés. En matière de fiscalité agricole, certains articles ont su faire consensus entre les deux chambres. Parmi ceux-ci, j'évoquerai la simplification des règles d'appréciation des produits des activités accessoires aux groupements agricoles d'exploitation en commun ou encore l'étalement sur cinq ans de l'imposition lorsqu'un agriculteur décide de passer de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés. Enfin, s'agissant de la transition énergétique, les deux chambres ont trouvé plusieurs points de consensus, en réduisant le taux de TVA à 5,5 % pour l'énergie solaire thermique ou bien en créant une réduction d'impôt au titre de la mise à disposition de vélos pour les salariés. Enfin, le Premier ministre a annoncé devant vous l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants au 1 janvier prochain. Cette mesure, que vous aviez votée sur l'initiative de votre commission des finances, nous permet d'engager le dialogue sur le rythme de la transition écologique et son financement. De la même manière, le Gouvernement a émis un avis favorable sur un certain nombre d'amendements adoptés sur l'initiative du Sénat, et que l'Assemblée nationale a ensuite confortés en nouvelle lecture. Parmi ceux-ci, j'évoquerai l'amendement de M. Antiste exonérant de TVA les locations de navires de grande plaisance de courte durée à partir de la Guadeloupe ou de la Martinique

plusieurs articles introduits par le Sénat dans la seconde partie du projet de loi de finances ont fait l'objet d'une adoption conforme. Je pense, par exemple, à l'annexe budgétaire relative au financement de la recherche, qui a été complétée sur l'initiative de Mme Darcos afin de rendre compte des montants consacrés à la recherche fondamentale sur la lutte contre le cancer pédiatrique. Votre assemblée a également adopté un amendement du président François Patriat qui élargit le document de politique transversale concernant la lutte contre la fraude fiscale aux fraudes de toutes natures, aussi bien fiscale que sociale. En rationalisant les nombreux rapports transmis au Parlement en la matière, cette disposition permettra au Gouvernement de mieux informer les citoyens sur les actions conduites dans le cadre de la lutte contre la fraude aux prélèvements obligatoires et sur les moyens qui y sont consacrés. Je terminerai en soulignant le travail du Sénat sur l'article 13 , qui fait suite à l'affaire des « CumEx Files », et qui a été adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement. Vous avez proposé l'introduction d'un nouveau dispositif fiscal permettant de contrer les montages effectués sur les dividendes, adopté à l'unanimité, sur l'initiative de la grande majorité des groupes composant votre assemblée. Ce dispositif introduit deux retenues à la source de 30 % : la première sur toutes les commissions versées à des non-résidents lors de la restitution du titre, en cas de schéma de « CumCum » interne la deuxième sur tous les paiements de dividendes vers des personnes résidant dans des États avec lesquels notre convention interdit à la France de prélever une retenue à la source, en cas de schéma de « CumCum » externe. Cette proposition a été partiellement modifiée par l'Assemblée nationale, tout en conservant l'esprit du dispositif initial, afin de se conformer au droit européen et aux conventions fiscales qui auraient pu le neutraliser. Je me réjouis d'autant plus de cette initiative qu'elle s'inscrit dans la continuité des objectifs du Gouvernement et de la majorité présidentielle pour lutter contre la fraude. Malgré certaines convergences que je viens d'exposer, la commission mixte paritaire a souligné des désaccords majeurs entre les deux chambres. les sénateurs, de vous faire part de l'incompréhension du Gouvernement face à certaines critiques qui ont été soulevées durant l'examen du projet de loi de finances en première lecture, votre assemblée ayant remis en cause les équilibres budgétaires, fiscaux et politiques de ce texte. Tandis que nous faisons le choix de mesures structurelles, le Sénat considère que nous menons une politique de « super-rabot », où nos seules économies- permettez-moi de reprendre vos mots, monsieur le rapporteur général -seraient engendrées par des « fusils budgétaires à un coup Ces mots contrastent pourtant avec l'ampleur des réformes engagées par le Gouvernement : réforme du travail et des politiques de l'emploi, réforme du logement et du financement du logement social, réforme de l'État et des services publics, réforme du recouvrement de l'impôt, réforme de l'audiovisuel public, ou encore réunion des réseaux de l'État à l'étranger. Je ne pense pas que l'on puisse qualifier de « méthodes de l'ancien monde » ces réformes qui ont vocation à transformer le fonctionnement de l'État en profondeur. Le deuxième point de désaccord majeur entre l'Assemblée nationale et le Sénat a trait et le Sénat a trait au financement des politiques publiques. Le rejet de six missions du budget général conduit à réduire fictivement les dépenses de 56,7 milliards d'euros. Le Sénat ne prévoit ainsi plus aucun crédit pour les missions « Cohésion des territoires », « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », « Écologie, développement et mobilité durables

des dépenses publiques. Vous vous engagez au mieux à les stabiliser, et toutes les réformes structurelles restent à accomplir. Elles seront encore plus difficiles à mener l'année prochaine et les années à venir, au moment où la croissance

de l'objectif initial. Au-delà de ces divergences fondamentales sur le contexte macroéconomique, nous regrettons que l'Assemblée nationale ait rétabli son texte

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2019 intervient dans un contexte nouveau, un « contexte bouleversé », pour reprendre les mots du rapporteur général, un contexte politique quasi insurrectionnel, à peine apaisé par les annonces du Président de la République.

Je l'ai dit à plusieurs reprises lors de nos discussions : nos institutions et nos corps intermédiaires doivent reprendre la main pour que notre pays sorte de cette crise par le haut. Le référendum d'initiative citoyenne est le nouvel avatar de cette défiance à l'égard de la démocratie représentative. Gaulliste libéral d'esprit, ... Ah ? ... je ne suis pas par principe hostile au référendum, bien au contraire. Mais il ne doit pas servir de prétexte à un nouvel antiparlementarisme. Nous refusons Nous refusons la tentation d'une tyrannie de la minorité, comme l'a dit récemment le président Gérard Larcher. L'urgence est aujourd'hui que les Français participent aux élections, qu'ils réinvestissent le champ démocratique en commençant par s'inscrire sur les listes électorales. On en est loin aujourd'hui C'est à nous, mes chers collègues, c'est à nous parlementaires, ici au Sénat et dans nos territoires, d'apporter des réponses à nos concitoyens. C'est au Gouvernement de proposer des solutions concrètes aux revendications légitimes qui se sont exprimées ces dernières semaines. Le Gouvernement gouverne, le Parlement légifère, dans le souci de l'intérêt général. Tel est l'esprit de nos institutions, et il doit être respecté. Or, le Sénat n'a pas à rougir de son rôle pendant la crise. Il a parfois, comme le rappelait M. le rapporteur général, anticipé la tournure des événements et proposé des mesures de bon sens. Je pense, bien sûr, au premier chef, au gel de la trajectoire carbone de la TICPE. Nous nous félicitons que l'Assemblée nationale ait adopté cette avancée politique du Sénat,

Nous étions convaincus que cette hausse était à la fois injuste, contre-productive et absolument pas écologique, puisqu'il n'existe pas d'alternative au GNR pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Nous nous félicitons donc de cette suppression, et ce d'autant plus que nous n'avions pas été suivis totalement par le Sénat sur ce point. Au total, ce sont 4 milliards d'euros de hausse prévue de la fiscalité écologique qui viendront à la place alimenter le pouvoir d'achat des ménages et le taux de marge des entreprises. C'est une bonne nouvelle pour nos concitoyens. C'est une preuve de lucidité du Gouvernement, qui doit beaucoup aux travaux du Sénat. Le contexte dans lequel nous examinons ce projet de loi de finances est également nouveau sur le fond. Il sert à présent de véhicule, avec le projet de loi que nous examinerons vendredi, aux mesures de pouvoir d'achat annoncées par le Président de la République. C'est notamment le cas de la nouvelle bonification de la prime d'activité avancée au 1 janvier 2019. C'est aussi le cas, malgré quelques hésitations, de l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires, du relèvement du barème kilométrique et du doublement de la prime à la conversion pour les « gros rouleurs ». Tout cela était indispensable. Néanmoins, sans préjuger des débats que nous aurons vendredi et sans nier la nécessité de ces mesures, nous nous interrogeons toujours sur les modalités pratiques de leur application, et surtout sur leur financement. Le Gouvernement a pris dans l'urgence les mesures qui s'imposaient. Il convient à présent de passer de la gestion de crise à la réforme structurelle. Le plus dur reste donc à faire. Le plus dur, c'est de réduire résolument la dépense publique et la masse salariale de l'État. Le plus dur, c'est de supprimer les dépenses publiques inefficientes et les niches fiscales poussiéreuses. Le plus dur, c'est d'avoir le courage de ne pas renoncer aux réformes vitales promises aux Français. Le plus dur, enfin, pour le Sénat, sera d'agir en responsabilité, sans critiques caricaturales, pour sortir le pays de l'ornière. La France ne peut plus se permettre un quinquennat pour rien. L'intérêt national commande un retour à la marche normale des institutions et au respect mutuel du Gouvernement et du Parlement. Mes chers collègues, nous sommes au bord du précipice, dans une situation quasi insurrectionnelle, et nous n'avons aucune raison de nous réjouir des difficultés que rencontre le Gouvernement. Je suis profondément convaincu que, si nous étions aux affaires, nous rencontrerions les mêmes difficultés,

de ces modifications qu'elles ont finalement débouché sur un effort inégalé depuis au moins dix ans en faveur du pouvoir d'achat des Français. J'entends bien sûr les critiques sur le déroulement de ce débat budgétaire. Toutefois, après toutes ces itérations,

que la France s'est mise à recréer de l'emploi dans le secteur privé et que le taux de chômage devrait passer sous les 9 % l'an prochain. C'est toujours trop, mais il faut remettre en perspective toutes les informations que nous avons reçues, notamment celles, récentes, de l'INSEE. figure notamment désormais l'accélération du versement de la prime d'activité que nous avons votée par amendement. Il existe dans notre pays trop d'actifs pauvres, nous savons

territoire par territoire, et de ce qui fonctionne en matière de mobilité, d'énergie, de déchets, de logement. Dans ce domaine, les collectivités locales, en lien avec l'État, font beaucoup. Si nous avons gelé la taxe carbone- le Sénat l'avait demandé, je l'ai déjà reconnu dans un

cette nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2019 s'apparente plus à une forme d'exercice imposé qu'à un véritable débat parlementaire. Alors que notre avenir commun se cherche et que s'impose un devoir d'innovation, nous demeurons- c'est le moins que l'on puisse dire -dans un carcan budgétaire et politique bien suranné. La commission mixte paritaire a en effet matérialisé son échec dans la production d'un rapport succinct et frustrant, qui laisse le Gouvernement à sa conviction d'avoir agi au mieux sur le chemin de la réduction des déficits. À la vérité, ce projet de loi est déjà caduc et déconnecté du bouillonnement de revendications et d'idées émergeant dans la société. Il conviendrait de le réécrire de fond en comble pour l'adapter à la situation concrète du pays et des Français. à l'irruption, lors de l'examen de ce projet de budget, d'une partie importante de la société, du monde du travail, des agents et des usagers des services publics, des chercheurs, des retraités, des assurés sociaux, des étudiants, des lycéens, des artisans, des salariés privés d'emploi, bref, d'une démocratie sociale. Tous disent, chacun avec ses mots : « Ça suffit ! », « Assez d'injustice sociale ! », « Assez d'injustice fiscale ! », « Le monde que vous nous promettez, celui d'un ruissellement qui ne viendra jamais, n'est pas le nôtre Oui, les Français commencent à envisager leurs activités sociales autrement que comme un coût et pointent les contradictions entre les sacrifices qu'on leur impose depuis des décennies et l'accumulation indécente de richesses. l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, la gabegie encouragée de l'évasion fiscale, la baisse de l'impôt sur les sociétés ou encore les facilités fiscales accordées aux actionnaires ne créaient ni l'emploi de demain, ni même celui d'après-demain. Ils dénoncent l'effacement dramatique des services publics et soulignent, avec nombre de leurs élus locaux, la folie que constitue le dogme de la baisse ininterrompue des dépenses publiques utiles- ces élus locaux que vous considérez non comme des « premiers de cordée », mais comme des « premiers de corvée ». Enfin, et c'est assez inédit, ces Français ne culpabilisent pas de réclamer leur dû sur leur fiche de paie et osent revendiquer une augmentation de leur pouvoir d'achat. Dois-je vous dire que notre groupe se sent « à l'aise dans ses baskets » et y voit toutes les raisons d'encourager un renforcement de la souveraineté populaire et de sa représentation, plutôt qu'un présidentialisme sans limites ? Dois-je rappeler, à l'aune de ces aspirations, notre groupe a contribué, avec ses amendements et ses votes, à leur traduction dans ce projet de loi de finances pour 2019 ? Pour nous, en effet, la logique des droits humains, économiques, sociaux, politiques ou culturels, collectifs ou individuels, doit primer sur la rentabilité financière et sur la prétendue domination idéologique de quelques-uns. C'est bien le sens des propositions transformatrices que nous aurions encore souhaité promouvoir en nouvelle lecture. Et nous en avons de nombreuses ! Pour baisser le coût de la vie de nos concitoyens tout en répondant à l'urgence climatique, à l'heure où la COP24 est loin de répondre à ce défi, ne vous contentez pas d'un chèque énergie, monsieur le secrétaire d'État, et mettez par exemple en place un plan d'urgence pour la rénovation des logements, qui sont de véritables passoires thermiques. Instaurez une baisse de la TVA sur les factures EDF et GDF, dont les tarifs n'arrêtent pas de flamber. Cessez de plomber les budgets des collectivités territoriales qui innovent et répondent aux besoins des populations, par exemple en finançant les cartes de transport des jeunes ou des précaires, voire en instaurant la gratuité de leurs transports collectifs. Avec quel argent ? Au lieu de cela, vous nous inventez des mesurettes, en décalage complet avec l'urgence sociale et qui ne changent rien à l'ornière dans laquelle nous enfonce votre politique. Vous épargnez soigneusement les plus fortunés. Vous refusez de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, d'élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu. Vous matraquez fiscalement les salariés, en repoussant notre proposition

est, s'agissant de la fiscalité des entreprises comme des prélèvements sociaux les concernant, vous renoncez à sortir de cette solidarité fiscale à l'envers, qui fait payer plus les petites entreprises et moins les entreprises les plus importantes. d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, du régime des groupes, de la consolidation des résultats, de l'optimisation du crédit d'impôt recherche, du suramortissement des équipements : toutes mesures qui auront surtout soutenu les profits et les dividendes. Ce sont ces groupes qui ont la main sur le magot des 165 milliards d'euros d'exonérations et dégrèvements accordés aux entreprises. Notre proposition de réforme fiscale vise clairement à inverser l'ordre des priorités et à combiner justice sociale et efficacité économique.

sur de nombreux points. Elle évite aussi au Gouvernement de s'expliquer sur ses choix, bien sagement assumés par sa majorité à l'Assemblée nationale, lesquels ne passeront pas sous le tapis

avec un niveau de TVA jamais atteint, des taxes sur les carburants de plus en plus lourdes, partagées pour financer des politiques sociales, et une fiscalité écologique qui commence à prendre du volume, utilisée qu'elle est en remplacement d'autres prélèvements fondés sur d'autres assiettes. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour examiner en nouvelle lecture le projet de loi de finances pour 2019, après une commission mixte paritaire non conclusive. l'occasion de constater une amorce de changement d'attitude du Gouvernement et de l'Assemblée nationale vis-à-vis des apports du Sénat. Encore quelques efforts, et la navette parlementaire rejouera parfaitement son rôle. Pour l'instant, malheureusement, quelques détricotages de nos textes persistent. Le meilleur exemple est celui de la lutte contre la fraude fiscale, à la suite du scandale des « CumEx », qui permet d'éviter l'imposition sur les dividendes, voire d'engranger des bénéfices indus Six groupes du Sénat, à la suite d'un travail de grande qualité conduit par notre commission des finances, ont déposé chacun un amendement visant à pallier les déficiences de la législation actuelle. Ces amendements ont fait l'objet d'un vote unanime, incluant les membres du groupe de la majorité présidentielle. Pour autant, le Gouvernement a fait le choix, en faisant proposer cette mesure par sa majorité à l'Assemblée nationale, de dénaturer complètement ce dispositif et, en pratique, de réduire sa portée contre des pratiques d'optimisation fiscale choquantes sur le plan éthique et coûteuses pour les finances de l'État. Ces demi-mesures permanentes sont incompréhensibles, aujourd'hui où s'exprime une demande forte de justice sociale. Elles témoignent à tout le moins d'un manque de considération du Parlement et de l'incapacité du Gouvernement à entendre les revendications des Françaises et des Français. Il n'y a qu'en matière de fiscalité environnementale, où le Sénat a voté à l'unanimité, quoique sans doute sur la base d'arguments différents selon les groupes, un amendement visant à supprimer l'augmentation des taxes sur le carburant, que le Gouvernement s'est finalement- et trop tardivement -rangé aux arguments de notre assemblée. Cette nouvelle lecture est aussi l'occasion d'évoquer le sort de plusieurs propositions qui ont été défendues durant les débats parlementaires par le groupe socialiste et républicain du Sénat, hier dénigrées, aujourd'hui reprises par le Gouvernement,

Nous avons estimé très tôt que l'élargissement de la « niche Copé » constituait un signal politique regrettable et accentuait une politique contribuant activement à des pratiques d'optimisation fiscale. Après avoir rejeté nos argumentations et notre amendement, le Gouvernement a fait marche arrière et a fini par entendre raison, à la suite d'un amendement déposé bien évidemment par sa majorité à l'Assemblée nationale.

Autre exemple : la semaine dernière, nous demandions qu'une partie du coût des mesures proposées par le Président de la République soit prise en charge par les très grandes entreprises de notre pays, sans que la majorité sénatoriale pipe mot. C'est chose faite pour les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour un montant de 1,8 milliard d'euros. Ce premier pas doit être poursuivi à l'avenir. Sur le sujet de la baisse de la taxation des entreprises, il faudra bien un jour mettre un terme à ce dumping fiscal, qui, de baisse en baisse et au nom d'une compétitivité toujours revendiquée, nous conduit inexorablement vers une taxation zéro à terme et à un transfert massif vers la taxation des revenus salariaux.

reste -et nous ne pouvons qu'être satisfaits de sa reprise, certes tardive, par le Gouvernement, sans attendre une éventuelle réglementation européenne, même si nous De la même manière- et bien que ce ne soit pas directement l'objet du présent projet de loi de finances -, je note que le Gouvernement a fait le choix de reprendre, au moins partiellement, plusieurs des propositions que les socialistes avaient déposées, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, en matière de pouvoir d'achat. Ainsi en est-il du relèvement à 2 000 euros du seuil pour l'augmentation de la CSG et de l'augmentation immédiate de la prime d'activité : autant de mesures, hier négligées, aujourd'hui partiellement, mais insuffisamment, mises en oeuvre. Il aura fallu une crise politique majeure pour que le Gouvernement ouvre enfin les yeux et revienne sur certaines des mesures annoncées en écoutant quelques-unes de nos propositions. Nous le regrettons, car cela discrédite globalement l'action publique et la vie politique dont nous avons collectivement la responsabilité. Il vous appartiendra, monsieur le secrétaire d'État, de veiller au respect de la parole donnée. nous avons encore quelques doutes sur ce point, mais vous serez jugé sur vos actes, c'est là le principe même de la démocratie. L'incroyable improvisation d'hier sur le chèque énergie- annulation le matin, réintégration l'après-midi -ne rassure pas sur ce point. Bien entendu, ce projet de loi de finances pour 2019 n'est plus en lien avec vos engagements en matière de trajectoire budgétaire. Nous notons que les mesures seront, pour une part significative, financées par des diminutions de dépenses sur des missions qu'il serait opportun, dans un souci de transparence, d'indiquer au plus vite. À ce titre, n'aurait-on pas pu demander plutôt un effort supplémentaire aux grands groupes ? L'année dernière, vous n'aviez pas hésité à prélever 5 milliards d'euros, et non 1,8 milliard d'euros comme aujourd'hui, au titre du remboursement de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés.

Nous notons enfin que vous ne traitez à aucun moment de la problématique de la justice fiscale, qui est pourtant l'un des piliers des revendications actuelles.

est indiscutablement à l'origine de ce sentiment d'injustice fiscale que vous n'hésitez pas vous-mêmes aujourd'hui à dénoncer, faisant de chacun de vous une espèce de pompier pyromane.

Un rééquilibrage de l'imposition en France est pourtant nécessaire pour rétablir un réel consentement à l'impôt. La question n'est pas tant celle du niveau des prélèvements obligatoires, ... Si ! ... qui servent- faut-il le rappeler en ces temps de doute sur le sens de l'action publique ? -à financer l'ensemble de nos services publics au bénéfice de tous, que celle de la juste contribution. L'impôt doit être réparti entre tous les citoyens « en raison de leurs facultés ». Cet extrait de l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prend aujourd'hui tout son sens. Chers collègues de la majorité sénatoriale, ... C'est la

nous sommes toujours fermement opposés à ce projet de loi de finances, malgré l'intégration partielle de plusieurs de nos suggestions. Je sais, monsieur le secrétaire d'État, selon le d'aujourd'hui, que ce n'est sans doute ni « subtil » ni « intelligent

entraînera le rejet du texte, est davantage dictée par des impératifs d'agenda, l'Assemblée nationale ayant elle-même achevé ses travaux vers six heures ce matin, que par des considérations strictement politiques. Mon groupe le regrette profondément, car, encore une fois, le Sénat ne pourra pas exercer jusqu'au bout ses prérogatives de législateur, dans le contexte social que nous connaissons. Il faudra tout de même un jour sérieusement s'interroger sur les conditions parfois ubuesques dans lesquelles le Parlement débat et vote la loi. Sauf à tout faire pour multiplier les malfaçons législatives, il n'est pas raisonnable que nous légiférions sur des sujets graves et sérieux à des heures aussi tardives. Chaque année, mon groupe ne peut que se désoler de ces conditions d'examen du projet de budget, qui nous obligent à survoler des sujets complexes tant par leur multiplicité que par leur technicité. Quoi qu'il en soit, après plus de 2 000 amendements déposés en première lecture et à nouveau 1 200 hier à l'Assemblée nationale, le Sénat devrait faire preuve d'une grande diligence, au milieu d'un ordre du jour sans cesse modifié. Nous ne pouvons non plus abstraire notre discussion d'aujourd'hui de l'examen, vendredi, du projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales. Je veux le redire la crise que traverse notre pays n'est pas qu'une simple saute d'humeur, elle est l'expression d'un mal plus profond, enkysté depuis plusieurs décennies, qui s'est développé au gré de gouvernements successifs. Le refus massif de la hausse des prix des carburants n'a été qu'un symbole et qu'un symptôme. Ce que beaucoup de nos concitoyens interrogent aujourd'hui, c'est bien notre pacte social. Bien sûr, l'ordre républicain a été rétabli après les dérapages et violences inacceptables qui ont connu leur paroxysme le 8 décembre dernier. Nous nous en réjouissons- je l'ai exprimé à plusieurs reprises -, même s'il ne s'agit que d'un préalable. L'intervention du Président de la République a apporté des réponses concrètes à l'urgence politique et sociale, même si les annonces doivent encore se transformer en actes. Je sais, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement veillera fermement à ce que les décisions du Président du Président de la République soient traduites dans la loi ! Oui, la loi est l'expression de la volonté générale et la haute administration n'en a certainement pas le monopole : la technocratie après le politique, et pas avant Finalement, ce projet de loi de finances a de fortes chances d'être modifié son encre à peine sèche. Le grand débat annoncé par le chef de l'État pour le début de l'année 2019 apportera son lot de propositions et d'innovations,

a été revu à la hausse de 0,1 point pour 2018 et, surtout, de 0,4 point pour 2019, repassant au-dessus de la barre des 3 C'est une inflexion importante, mais nécessaire, pour répondre à l'urgence économique et sociale, même si le rétablissement des finances publiques doit rester un outil du développement de notre pays. Comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas non plus ignorer le contexte européen. Aux incertitudes politiques que nous connaissions- coalition populiste en Italie, Brexit au Royaume-Uni -s'en ajoutent d'autres, comme la chute du gouvernement belge hier sur la question migratoire. L'Europe et, plus largement, nos démocraties occidentales sont atteintes de convulsions inquiétantes. Notre modèle politique et social est lui-même remis en cause. Notre débat budgétaire en subit les conséquences, quand bien même il ne s'agit que d'une question secondaire au vu des tensions que nous traversons. Plus modestement, le Sénat a également connu son lot de tensions, avec les sautes d'humeur des uns ou des autres. Toutefois, gardons le sens de la mesure. Dans le contexte actuel, cet épisode doit surtout nous appeler collectivement, Gouvernement et majorité sénatoriale, à la responsabilité. Nous incarnons la démocratie représentative et sommes, à ce titre, tenus d'agir pour l'intérêt général, corollaire de la confiance placée en nous par nos concitoyens. Certes, cette confiance varie dans le temps, allant même jusqu'au rejet des institutions. Néanmoins, rien ne serait pire que de diluer les corps intermédiaires, au premier rang desquels les élus et les maires, piliers de la République. Très attaché au rôle du Parlement, mon groupe regrette- sans naïveté, rassurez-vous ! -que l'Assemblée nationale et le Sénat n'aient pu parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Je me félicite toutefois de la reprise de certains de nos amendements par les députés, parmi lesquels le maintien de la taxe sur les friches commerciales le rétablissement du régime fiscal des sociétés d'intérêt collectif. Enfin, nous nous félicitons qu'aboutisse notre combat historique pour le plafonnement de l'exonération d'impôt sur les hauts revenus de journalistes, rédacteurs et critiques Nous avions encore une fois raison trop tôt et je me réjouis que les députés aient rejoint les sénateurs pour supprimer cet avantage injustifié. En revanche, je regrette naturellement que certains autres de nos amendements n'aient pas été retenus par l'Assemblée nationale. Je pense en particulier à la méthanisation des déchets,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues,

et de considérer que, si nous avions été mieux entendus, notamment sur le niveau exagéré des taxes et sur le diesel, la situation de la France et de nos concitoyens serait bien meilleure, et ce à moindre coût. Aujourd'hui, un certain nombre de décisions nous sont proposées en urgence. Il y a fort à parier qu'elles ne satisferont pas tous nos concitoyens, ce qui est normal compte tenu de l'hétérogénéité des demandes. En outre, un certain nombre de mesures que nul n'avait réclamées sont maintenant

je vous propose une solution qui aurait pour avantage de ne pas déséquilibrer nos finances tout en créant de la confiance. Car ne vous y trompez pas, mes chers collègues, les Français ne sont pas dupes et n'ont pas envie qu'on les roule une fois de plus dans la farine La suppression de la taxe d'habitation est une mauvaise chose, car elle est injuste financièrement. Elle n'apporte aucun pouvoir d'achat supplémentaire à ceux qui ne la paient pas.

votre temps de parole ! ... s'agissant du grand débat qui est proposé aux Français. Nous savons d'expérience que la confusion des idées est propice à l'instrumentalisation. Il s'agit alors d'atteindre des objectifs qui n'ont rien à voir avec les souhaits profonds exprimés par certains de nos concitoyens.

en débattre. Vendredi, nous allons voter d'autres mesures, dont l'impact financier aurait peut-être pu être prévu dans l'ensemble, mais tant pis ... Monsieur le secrétaire d'État, c'est dommage, franchement, que cela tombe

la responsabilité de vous dire : nous sauvons le Gouvernement, nous faisons en sorte que la parole du Président de la République- non pas Emmanuel Macron, mais le Président de la République de la V République -ait encore du sens. C'est cela la France

Cette « double année », si l'on peut dire, car elle verra l'apurement de la dette de l'État envers les entreprises au titre de l'exercice 2018 et le financement des allégements de charges dès le mois de janvier 2019, représente un effort de 0,9 point de PIB. Cela nous amène à considérer

Quant à l'atténuation de la trajectoire de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros, elle sera proposée au Parlement, et donc à votre assemblée, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Nous gardons en

La discussion générale est close. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Ils ne trouvent pas une combine une prime d'activité : ils assument. Ils savent ce que c'est qu'une rémunération ; ils savent ce que c'est qu'un salaire. Et ils ont décidé de l'augmenter de 22 %.

Ce n'est pas une menace ! Vous verrez dans les comptes de l'État ce que coûtera cette décision ; celle-ci, en effet, impacte les classes moyennes de ladite « outre-mer », qui sont des pourvoyeuses de pouvoir d'achat.

agios bancaires, services bancaires, taux d'intérêt, etc.- je ne parle même pas de l'alimentation, qui relève du minimum quotidien obligatoire. Vous verrez les conséquences

maintenant le verdict : notre groupe va s'abstenir sur cette motion tendant à opposer la question préalable. Nous sommes bien d'accord que, dans un tel

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande Le scrutin est ouvert.

2019 est rejeté. Je n'ai été saisie d'aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents. Elles sont donc adoptées.